au CSA ? Le CSA est une autorité administrative qui, dans un premier temps, a été chargée d'attribuer des fréquences radio

afin que des personnes, des usagers qui ne veulent plus utiliser les réseaux sociaux, puissent faire migrer librement leurs données vers d'autres plateformes, et d'un point essentiel, qui permettra également de conforter la liberté d'expression. Si, d'aventure, on s'apercevait que les réseaux sociaux mettent en place des systèmes pour brider l'information

jouant un rôle particulier dans la diffusion et la propagation des contenus haineux, le présent amendement tend à inclure les moteurs de recherche dans le champ des opérateurs concernés par la nouvelle régulation des plateformes, qui seront désormais assujettis à des obligations de moyens renforcées, sous la supervision du CSA. À l'instar des opérateurs de plateformes en ligne, les moteurs de recherche exercent un rôle d'intermédiaires actifs permettant le partage de contenus

dans son avis sur la présente proposition de loi en vue de respecter le principe constitutionnel d'égalité et le principe conventionnel de non-discrimination.

plus aucun hébergeur ne serait soumis à la régulation et aux obligations de moyens sous la supervision du CSA. Nous y sommes donc défavorables. L'amendement n° 43 de M. Montaugé vise à réintroduire les moteurs de recherche dans le champ des opérateurs supervisés par le CSA.

licite. Pour entrer dans le détail, monsieur Montaugé, les moteurs de recherche, dans leur fonctionnement technique, leur finalité et leur effet sur la viralité d'un contenu, se distinguent substantiellement des réseaux sociaux. des réseaux sociaux. Ils organisent la visibilité des contenus sur le net de façon algorithmique, constante et prévisible. Il n'y a normalement aucun traitement particulier en fonction de l'identité de l'auteur de la recherche.

Les moteurs de recherche ne contribuent pas, comme le font les réseaux sociaux, à la viralité d'un contenu. L'utilisateur d'un moteur de recherche n'y voit que les informations qu'il est venu chercher en fonction de sa requête, contrairement aux réseaux sociaux sur lesquels une foule de contenus publiés par ses contacts lui sont proposés. Si les moteurs de recherche contribuent à la visibilité des sites internet, ce ne sont pas eux qui rendent directement ces sites ou les contenus publics. Un site se retrouve référencé dans le moteur de recherche, non pas à la demande de son auteur, mais automatiquement. automatiquement. Enfin, les moteurs de recherche ne stockent pas les contenus, ils les référencent. Ils ne peuvent pas bénéficier techniquement du recours à certaines bases de données de contenus illicites. je l'ai dit, les caractéristiques techniques des moteurs de recherche rendent quasiment impossible de désindexer un seul propos haineux sans rendre inaccessible tout le reste d'une page ou d'un site pourtant licite. Un passage haineux peut être présent sur un site indexé à côté de bien d'autres passages qui ne le sont pas. par exemple, à un commentaire sur la page d'un média, d'un forum ou d'un site consacré à des débats participatifs : faut-il pour autant déréférencer le site entier au risque d'atténuer significativement sa visibilité sur internet et la liberté d'expression des autres utilisateurs ? Pour conclure, je note que la loi allemande, la ,les

a une expérience certaine en matière de contenus, notamment à la télévision. Il est évident que les usages et les pratiques des Français évoluant, la compétence du CSA doit s'étendre au numérique. Il est normal qu'il s'adapte aux usages du temps. Cela représente un défi

qui n'est pas mis en évidence, alors qu'il me semble justifier le maintien de cet amendement : les moteurs de recherche et leurs algorithmes renvoient à chaque internaute

mon point de vue, on doit favoriser l'émergence de solutions alternatives, non pas pour permettre à ceux qui répandent des propos haineux de le faire ailleurs, mais tout simplement pour laisser le choix à celles et ceux qui refusent d'utiliser les réseaux sociaux actuels pour des raisons éthiques de faire migrer leurs données sur d'autres réseaux beaucoup plus transparents, utilisant des algorithmes qui répondent à un code moral

J'ai lu dans un article la semaine dernière que Twitter finançait une petite équipe indépendante comptant jusqu'à cinq architectes, ingénieurs et designers open source pour développer des normes ouvertes et décentralisées pour les médias sociaux, l'objectif étant que Twitter soit finalement un client de cette plateforme.

Autant il ne me semble pas possible d'inscrire le délai de vingt-quatre heures à l'article 1 comme objectif de résultat, autant en faire une obligation de moyens est une piste intéressante. Cette rédaction tente en effet de rester sur la ligne de crête. Elle me semble compatible avec le droit européen, puisqu'elle ne fixe ni délai couperet ni obligation de résultat exhaustif pour tous les types de contenus à laquelle on ne peut déroger et sous la menace de sanctions pénales. Elle fixe, en revanche, une obligation de moyens, un objectif de délai, un principe, une moyenne à observer, sauf circonstances exceptionnelles : afflux massif de signalements difficiles à évaluer, pannes imprévisibles, etc. Cette rédaction inscrit « en dur » dans la loi la durée de vingt-quatre heures. Elle liera bien les plateformes qui devront en tenir compte et elle servira d'indication au CSA pour son contrôle périodique. Le régulateur pourra en assurer le respect en cas de dépassement injustifié, si les plateformes ne se dotent pas des moyens d'atteindre cet objectif

ou non du contenu publié en ligne entre son auteur et la plateforme où le contenu a été publié. Actuellement, la loi du 22 décembre 2018 prévoit que, lorsque l'auteur du contenu est en désaccord avec la notification, celui-ci reste en ligne jusqu'à ce qu'un juge tranche. Cela vise à faire primer la liberté d'expression sur la censure. L'article 2 inverse ce principe, en prévoyant que, dorénavant, en cas de litige, le contenu sera supprimé ou rendu inaccessible. Or nous ne disposons pas d'étude d'impact pour évaluer les risques sur la liberté d'expression. En outre, nous ne sommes pas à même de juger si ces situations conflictuelles sont fréquentes et nous ne connaissons pas la politique des plateformes dans ces cas-là. Le seul retour d'expérience dont nous disposons nous vient d'Allemagne, où près d'un million de notifications ont eu lieu en un an, donnant lieu à la suppression des contenus dans 17 % des cas. Ces chiffres peuvent être interprétés différemment : ils signifient soit que les utilisateurs ne connaissent pas bien la loi allemande et sur-notifient, soit que les plateformes ont une politique très libérale de maintien des contenus notifiés. En l'absence de données plus précises, il nous paraît pertinent d'adopter une attitude prudente de maintien du droit existant plutôt que de mettre en place un système de notification qui pourrait aboutir à un outil de censure puissant.

tend à prévoir une voie de recours quand l'usager considère que ses messages ont été censurés à tort.

En l'espèce, en cas de contre-notification par l'auteur de contenus litigieux retirés, la plateforme devrait obligatoirement les rétablir, à charge pour le notifiant de saisir le juge des référés. Même si je suis favorable sur le principe à la démarche,

part, concernant l'intérêt pour agir du requérant, une notification de contenu haineux ou illicite à un hébergeur peut émaner de toute personne, sans qu'elle ait à justifier être personnellement lésée par ledit contenu. Or, devant le juge, son action devra bien s'appuyer sur un tel intérêt, sauf à permettre une sorte d'action populaire. D'autre l'articulation avec le régime de responsabilité de la LCEN, le dispositif envisagé oblige la plateforme à rétablir certains contenus litigieux dans l'attente de la décision du juge, laquelle peut prendre une semaine et lui donner tort, alors même que la plateforme engage sa responsabilité pénale et civile si elle ne les a pas retirés

retirés. Bien entendu, nous avons lu avec attention les observations de la Commission européenne relatives au risque de surveillance générale. Nous ne sommes pas dans ce cas. D'une part, il s'agit d'une obligation de moyens. C'est la raison pour laquelle nous avons mentionné que les moyens mis en oeuvre par la plateforme sont des moyens « appropriés part, comme en droit interne, le droit européen est sujet à interprétation lorsqu'il est question de l'appliquer. À ce propos, la Cour de justice de l'Union européenne a eu à se prononcer le 3 octobre dernier, dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation des articles 14 et 15 de la directive e-commerce, afin de savoir si l'obligation de retrait de certaines informations illicites imposée à un hébergeur vise également d'autres informations identiques. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, la directive e-commerce du 8 juin 2000 ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction d'un État membre puisse enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu'il stocke et dont le contenu est identique à celui d'une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l'accès à celles-ci, quel que soit l'auteur de la demande de stockage de ces informations, dès lors qu'une telle injonction est limitée à des informations véhiculant un message dont le contenu demeure, en substance, inchangé par rapport à celui qui a donné lieu au constat d'illicéité, et qu'elle comporte les éléments spécifiés dans la demande. En outre, il faut qu'une telle opération ne soit pas de nature à contraindre l'hébergeur à procéder à une appréciation autonome de ce contenu. Dans ce cadre de l'Union européenne, il est nécessaire de prévoir que les opérateurs mettent en oeuvre les moyens appropriés pour empêcher la rediffusion en ligne de contenus illicites identiques.

J'ai bien suivi votre raisonnement, monsieur Montaugé : vous voulez rétablir cette obligation générale d'empêcher la réapparition des contenus illicites, le principe, qui est contraire

M. David Assouline, pour explication de vote.

dans cette loi aussi, vous aviez prévu la nomination d'un représentant. Or ce dispositif n'a pas fonctionné. Vous le remplacez aujourd'hui par la notion de « point de contact Expliquez-nous ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce une paillote dans un coin du territoire où l'on vient pour essayer de rencontrer M. Google ou M. Twitter ? Je ne vois pas, d'un

parfaitement ne pas répondre à la convocation de la justice française. Je doute que leur imposer un point de contact puisse résoudre ce problème.

substitution qui tend aussi à répondre à de possibles réserves en provenance de la Commission européenne, l'obligation d'un représentant légal sur le territoire français pouvant être possiblement considérée comme une entrave injustifiée au principe de la libre prestation des services de la société de l'information dans le marché unique.

parce que vous avez mal ficelé ce texte, il apparaît qu'il n'est pas possible de lutter contre les contenus haineux

Or, à une époque où une part croissante de nos concitoyens a recours aux réseaux sociaux et aux plateformes en ligne pour accéder à de l'information, la prolifération des faux comptes, créés uniquement à des fins de dissémination d'informations douteuses et parfois même haineuses, constitue une menace majeure pour la liberté d'expression et la bonne information des citoyens. Ce texte ne saurait ignorer cet aspect du problème. Cet amendement vise donc à faciliter la lutte contre ces faux comptes. Il crée, pour cela, une obligation de moyens à destination des plateformes, afin que celles-ci se dotent des capacités de ciblage et de suppression des comptes que l'on soupçonne être des faux, utilisés pour répandre des contenus haineux. Pour cela, nous proposons de retenir la technique du faisceau d'indices, qui, malgré son origine prétorienne, s'applique d'ores et déjà dans le domaine des marchés publics. Afin de ne pas porter atteinte aux équilibres du texte, ces suppressions de comptes pourraient donner lieu à des réclamations similaires à celles qui sont prévues à l'article 2

rapporteure pour avis. Cet article constituera probablement l'héritage le plus durable et utile de la proposition de loi, puisqu'il pose les bases d'une régulation des acteurs du numérique menée par un CSA dont le champ de compétences sera significativement étendu par la future loi sur l'audiovisuel. Comme je le signalais dans mon propos introductif, nous sommes favorables à cette régulation, dont on parle depuis un certain temps d'ailleurs, et nous pensons que le CSA, qui du Parlement dans les mois qui viennent, est le plus à même d'accomplir cette mission. Je tiens à souligner que le texte que nous examinons ne confie à aucun moment au CSA la responsabilité de juger du caractère licite ou non des Sa mission est bien de s'assurer des moyens mis en oeuvre et de l'efficacité dans l'application des règles fixées par la loi. Je formulerai trois autres observations. Premièrement, je remercie la commission des lois d'avoir réservé une suite favorable aux amendements de la commission de la culture. Nous avons simplement cherché à mieux encadrer l'intervention du régulateur et je crois que le texte est meilleur sur ce point.

-s'intéresse actuellement de très près au projet de Facebook de fusion des infrastructures techniques du réseau social avec WhatsApp et Instagram. Des politiques militent aujourd'hui pour une application très stricte du droit de la concurrence aux géants du numérique, à l'instar de ce qui a été fait avec la Standard Oil

désignent un représentant légal exerçant les fonctions d'interlocuteur référent ». Si j'ai bien compris votre analyse, cet article pourrait aujourd'hui être anticonstitutionnel. Vous ouvrez la voie à

Aujourd'hui, ce sont elles qui jouent le rôle de chambre d'écho, ce sont elles qui amplifient les phénomènes que nous combattons ce soir.

pour prévoir le cas d'opérateurs ne réalisant pas de chiffre d'affaires ou réalisant un chiffre d'affaires temporairement ou artificiellement faible. Le fait de combiner un montant forfaitaire forfaitaire et un pourcentage du chiffre d'affaires permettra d'éviter des comportements opportunistes non prévus par le mécanisme actuel et d'aligner les sanctions sur celles qui sont prévues par le RGPD en matière de violation de données personnelles. La commission émet

proposition de loi a vocation, notamment parce qu'elle est extrêmement lourde à assumer, à ne s'appliquer qu'aux très grands réseaux sociaux.

émet un avis défavorable sur cet amendement, qui vise à attribuer au seul juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le contentieux des décisions de régulation des plateformes prises par le CSA. C'est une complexité inutile. Le droit commun de la compétence contentieuse a vocation à s'appliquer, faute de dérogation expresse par le législateur. Pour mémoire, le Conseil d'État est juge des recours dirigés contre les décisions prises par les autorités indépendantes au titre de leur mission de contrôle ou de régulation.

La création de mécanismes garantissant la lutte contre la duplication de contenus haineux doit être en effet au coeur du dispositif de lutte contre les contenus haineux. La mise en place d'un mécanisme de partage d'informations entre opérateurs renforcera la coopération systémique visant à lutter contre la haine sur internet. Le CSA pourrait organiser la coopération entre les plateformes pour éviter que des contenus rendus inaccessibles sur une plateforme ne restent disponibles sur une autre plateforme. Ce partage d'informations permettrait une réaction proactive des plateformes, dont le signalement de contenus illicites, et une lutte efficace contre les sites miroirs. par des plateformes et des moteurs de recherche dits « alternatifs », tend à permettre au CSA d'organiser un partage transparent d'informations entre tous les opérateurs, quelles que soient leur taille et leurs relations concurrentielles.

en place par la présente proposition de loi d'un mécanisme de coopération et de partage d'informations entre opérateurs est essentielle pour mieux lutter contre les contenus haineux sur internet, comme je viens de l'expliquer à l'instant. Il est tout aussi essentiel que le régulateur puisse organiser cette coopération et éviter que des contenus rendus inaccessibles sur une plateforme ne restent disponibles sur une autre plateforme, à qui ces contenus n'auraient pas été notifiés. Le régulateur doit être en mesure de fixer les principes et les modalités de mise en oeuvre des outils de coopération et de partage d'informations entre opérateurs.

la chance ! Tous ces amendements visent à préciser les modalités des échanges d'informations entre plateformes. Permettez-moi de rappeler quelques éléments de contexte. Alors que nos gouvernements renforcent les devoirs de coopération des plateformes, la constitution par les grands acteurs du numérique de base de données de textes et d'images illicites est une source d'efficacité notable dans leur lutte contre ces contenus. Des outils techniques leur permettent, par exemple, de comparer, de filtrer et d'éliminer de façon quasi automatisée les images illicites. Ils épargnent ainsi à leurs modérateurs humains une tâche difficile et font disparaître des contenus illicites avant même que leurs utilisateurs n'aient eu besoin de les leur notifier. Mais ces bases de données de contenus illicites constituent aussi désormais un enjeu économique majeur. Leur maîtrise est un moyen de conserver ou de créer de solides barrières à l'entrée, aux dépens de plateformes plus modestes. Je vous rappelle que, sur l'initiative de notre collègue rapporteur pour avis, Yves Bouloux, la commission des lois a précisé les missions confiées au CSA afin d'encourager le partage d'informations entre opérateurs. Les auteurs des trois amendements identiques n 8 rectifié, 38 et 50 rectifié souhaitent aller plus loin et imposer la mise à disposition de ces informations de façon gratuite. Malheureusement, en raison de la valeur économique des informations collectées par les plateformes, il me semble difficile d'adopter de tels amendements : ils s'apparentent à une forme d'expropriation sans prévoir de garanties ou d'indemnisation appropriée. Telles sont les raisons En revanche, la seconde partie de ces amendements, qui est reprise dans l'amendement de repli n° 39, me semble intéressante, et j'y suis favorable : il s'agit de donner au CSA compétence pour préciser le format de ces informations afin d'en faciliter la circulation entre plateformes, dans un format ouvert et conforme à ses recommandations.

En l'espèce, il n'apparaît pas évident que le CSA puisse imposer de tels standards de manière large à des acteurs non basés en France. Cette disposition pourrait en outre renforcer les interrogations soulevées par la Commission européenne sur le caractère ciblé et proportionné du dispositif, qui l'a conduite à poser des questions sur la conventionnalité de la loi. Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cette disposition. ? La commission des lois a souhaité, je le rappelle, donner au CSA la nouvelle mission d'encourager l'interopérabilité entre plateformes, afin de permettre aux victimes de haine de se « réfugier » sur des réseaux sociaux ayant des politiques de modération différentes, tout en tout en continuant à échanger avec les contacts qu'elles avaient noués jusqu'alors. Il s'agit ni plus ni moins d'approfondir l'obligation de portabilité en complétant la boîte à outils du régulateur des plateformes, conformément d'ailleurs aux recommandations de la commission d'enquête du Sénat sur la souveraineté numérique, dont

aux travaux en cours de la commission des affaires économiques et à la proposition de loi de notre collègue Sophie Primas visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace.

opportuniste de l'argument européen. Vous nous avez expliqué au début de ce débat que l'avis de la Commission européenne ne nous engageait pas et que la France devait montrer le chemin.

L'auditabilité et la redevabilité, au sens de « rendre compte », des algorithmes utilisés par les plateformes doivent être des objectifs du législateur. C'est l'une des recommandations de la commission d'enquête sénatoriale sur la souveraineté numérique. Cela suppose que les autorités concernées, dont les régulateurs, puissent avoir recours à une expertise spécialisée pour développer et mettre en oeuvre des techniques de contrôle adaptées. Sur ce point particulier, monsieur le secrétaire d'État, nous suivrons avec attention le projet de loi sur l'audiovisuel, qui prévoit, dans son article 36, la création d'un « pôle d'expertise numérique », lequel apporterait une expertise technique spécialisée aux autorités intervenant dans la régulation des opérateurs de plateforme en ligne,

ce pôle de travailler. Pour assumer les missions de régulation et de contrôle qui lui sont conférées par la présente proposition de loi, le CSA doit être en mesure, d'une part, d'évaluer et de garantir la transparence des algorithmes utilisés par les plateformes et, d'autre part, de vérifier leur conformité à la loi. L'alinéa 17 de l'article 4 de la proposition de loi prévoit que le CSA doit pouvoir obtenir auprès des opérateurs de plateformes en ligne « toutes les informations nécessaires au contrôle des obligations » prévues par la proposition de loi.

Cet amendement est intéressant, monsieur Montaugé, car il vise à préciser les pouvoirs de contrôle dont dispose le CSA pour assurer le respect des nouvelles obligations à la charge des plateformes en matière de lutte contre la haine. Ces pouvoirs figurent déjà dans la loi relative Il s'agirait, en l'espèce, de permettre expressément l'accès du régulateur aux systèmes algorithmiques utilisés par les plateformes, afin de pouvoir les auditer.

Nous proposons donc de réintroduire le dispositif de lutte contre les sites miroirs. Compte tenu des critiques qui ont été formulées par la commission des lois, nous sommes revenus sur la rédaction pour définir de manière exacte et, nous semble-t-il, appropriée les prérogatives de l'autorité administrative : cibler correctement les acteurs concernés, en excluant notamment les fournisseurs de noms de domaine, et en précisant que le blocage ou le déréférencement portent bien sur des sites, et non sur des

qui est souvent utilisée pour contourner un blocage. Ainsi, l'autorité administrative demandera aux opérateurs de plateformes, fournisseurs de noms de domaine et moteurs de recherche ou annuaires de retirer ou déréférencer, le cas échéant, des contenus relevant du champ d'application de la nouvelle loi dont la reprise totale ou partielle a été précédemment interdite par décision judiciaire passée en force de chose jugée. Lorsque l'opérateur ne se conforme pas à la demande administrative de retrait ou de déréférencement, l'autorité judiciaire peut être saisie en référé ou sur requête pour ordonner toutes mesures destinées à faire cesser l'accès à ces contenus. Nous avons déjà entamé ce débat en présentant notre amendement n° 44 à l'article 2 de la proposition de loi. proposition de loi. Le législateur connaît déjà bien ce problème, qui perturbe gravement l'efficacité des mesures de retrait. Actuellement, s'il existe plusieurs possibilités de blocage de contenus illicites sur internet, il n'est pas prévu de droit de suite lorsque les mêmes contenus haineux réapparaissent. Ces derniers sont considérés comme des contenus distincts et leur retrait exige d'enclencher une nouvelle procédure judiciaire pour obtenir le blocage alors que le nouveau site reprend à l'identique ces contenus.

ne s'oppose pas à ce qu'une juridiction d'un État membre puisse enjoindre à un hébergeur de supprimer les informations qu'il stocke et dont le contenu est identique à celui d'une information déclarée illicite précédemment ou de bloquer l'accès à celle-ci, quel que soit l'auteur de la demande de stockage de ces informations. Nous sommes précisément dans ce cas, l'autorité administrative agissant dès lors qu'elle a été habilitée à le faire dans la décision judiciaire. Enfin, nous avons veillé

l'annonceur publicitaire un compte rendu de la liste des domaines et sous-domaines sur lesquels l'annonceur a diffusé des publicités. En outre, un commissaire aux comptes doit attester que l'annonceur publicitaire est en possession de cette liste. le dispositif proposé est déjà en place et n'a pas besoin de faire l'objet d'une nouvelle disposition. En effet, le décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale prévoit déjà que le compte rendu communiqué par le vendeur d'espace publicitaire à l'annonceur précise la date et les emplacements de diffusion des annonces, ainsi que le prix global de la campagne et le prix unitaire des espaces publicitaires facturés. En outre, le dispositif proposé part d'un postulat erroné. En effet, la fourniture d'une liste de sites n'a d'intérêt que si ces sites sont illicites. aucun annonceur soucieux de sa réputation ne souhaite diffuser des publicités sur des sites haineux, car cela risque de porter atteinte à sa marque alors qu'il consent des investissements importants pour la valoriser.

Nous pouvons les partager. Cependant, l'amendement n° 47 de notre collègue Thani Mohamed Soilihi et des membres du groupe La République En Marche y répond avec un dispositif permettant d'agir sur le financement

Lors de l'examen en commission, le rapporteur a bien voulu considérer notre rédaction d'appel visant à tarir la source du financement de sites faisant commerce de leur haine en ligne en faisant jouer le dommage réputationnel pour les annonceurs publicitaires. La disposition ainsi adoptée l'article 6 AA vise à prévoir qu'un commissaire aux comptes atteste que l'annonceur publicitaire est bien en possession de la liste des domaines et sous-domaines internet sur lesquels le vendeur d'espaces publicitaires a diffusé des publicités. En cas de manquement de l'annonceur à cette obligation, l'autorité administrative pourrait prononcer une sanction pécuniaire ne pouvant pas excéder 4 % du chiffre d'affaires. L'amendement que nous présentons en séance vise à

Il prévoit ainsi que les annonceurs publient en ligne et tiennent à jour, au minimum mensuellement, les informations relatives aux emplacements de diffusion de leurs annonces qui leur sont communiquées par des vendeurs d'espace publicitaire. En cas de manquement à cette obligation, une amende administrative de 30 000 euros est prévue sous le contrôle des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le sous-amendement n° 63, présenté par

Costes. Le phénomène est à présent bien connu : la publication de contenus clivants attire davantage les utilisateurs de plateformes en ligne que celle de contenus modérés. Or le modèle économique des plateformes et des sites en ligne s'articule souvent autour de la location d'espaces publicitaires dont les revenus sont établis en fonction du nombre de fréquentations. Cela peut donc entraîner ces plateformes ou sites à promouvoir des contenus clivants potentiellement illicites pour s'assurer une fréquentation, donc des revenus minimaux. L'objectif de l'article 6 AA et de l'amendement n° 47, qui tend à le réécrire, est de lutter contre ce biais en renforçant la transparence sur toute la chaîne de publicité en ligne. Le sous-amendement que nous proposons s'inscrit dans le même esprit, en se concentrant sur les sites d'information, qui, eux aussi, se financent en partie par la publicité. Compte tenu de l'importance de ces sites pour le débat public, nous proposons de rendre obligatoire la publication d'un lien sur leur site, afin de permettre au lecteur de s'informer sur les sources de financement publicitaire de ces sites d'information.

dans le cadre du contrôle judiciaire ou de la mise à l'épreuve. Il s'agit, dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, de l'interdiction pour l'intéressé d'adresser des messages à la victime, de manière directe ou indirecte, par tout moyen, y compris par voie électronique.

prévoit la possibilité pour le juge d'enjoindre à l'intéressé de s'abstenir « d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction

du Gouvernement ? Le Gouvernement est défavorable à la suppression de ces dispositions, qui complètent selon nous tout à fait utilement la proposition de loi. Il est tout à fait opportun d'instituer dans le cadre du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, qui deviendra sursis probatoire au mois de mars 2020 en l'application de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice, une nouvelle interdiction, celle d'adresser des messages à la victime, notamment par voie électronique. Cela constitue notamment une réponse particulièrement appropriée aux faits de cyberharcèlement. Une telle interdiction est plus précise et plus ciblée que l'interdiction générale d'entrer en relation avec la victime, prévue par le 9° de l'article 138 du code de procédure pénale et le 13° de l'article 132-45 du code pénal. Il est en effet primordial que les personnes astreintes à une interdiction d'entrer en relation avec la victime dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve puissent percevoir la pleine portée des obligations et interdictions qui leur sont applicables. Il convient de rappeler que le non-respect d'une interdiction du contrôle judiciaire peut entraîner le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen et que le non-respect d'une interdiction prévue dans le cadre d'une mise à l'épreuve peut conduire à l'incarcération d'un condamné. Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de ces clarifications particulièrement utiles.

Sans remettre en cause l'importance du sujet, la création d'une nouvelle instance chargée du suivi de ces questions ne nous paraît pas pertinente. En effet, il nous semble au contraire qu'en parallèle de la vigilance du Parlement sur ces questions, il importe que le suivi soit assuré par les autorités de régulation elles-mêmes sans qu'il soit besoin d'institutionnaliser cette démarche. Cela relève simplement de la bonne administration. Je rappelle que notre vie républicaine est hantée de millefeuilles composés de nombreux observatoires, comités ou commissions dont l'effet sur la vie de nos concitoyens a été faible, voire parfois nul. Dans cet esprit, nous proposons de rendre plus effective la communication entre les autorités de régulation concernées entre elles et avec les différents acteurs du milieu.

Ainsi, de nombreuses images de policiers et de gendarmes ont été diffusées sur les réseaux sociaux, ce qui les rend facilement identifiables et en fait potentiellement des cibles, de même que leur famille. Ces diffusions ont bien souvent été accompagnées d'injures, d'appels à la violence et de menaces. Sauf dans certaines circonstances particulières, les membres des forces de l'ordre ne peuvent pas s'opposer à l'enregistrement de leur image lorsqu'ils effectuent une mission ni à sa diffusion. Or la préservation de leur anonymat garantit leur efficacité, mais aussi leur sécurité. Afin d'évaluer les conséquences de la diffusion de contenus haineux sur internet visant les forces de l'ordre, cet amendement de notre collègue Jean-Pierre Grand prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport

ne serait-ce qu'en raison de l'agenda européen très chargé, qui nous contraindra probablement à prendre de nouvelles mesures de transposition. Ce sera, je l'espère, l'occasion de travailler de nouveau

et de retours d'expérience plus nombreux, notamment de l'évaluation de la mise en oeuvre de la loi allemande. À ce stade, une majorité du groupe du RDSE votera pour ce texte, tel qu'il a été modifié par le Sénat. Les éléments les plus problématiques au regard de l'obligation de conformité au droit européen ont été retirés. Il ne reste finalement presque que du « droit mou » : l'extension du pouvoir de recommandation du CSA et la création d'un observatoire qui lui serait rattaché. Finalement, après les travaux de notre assemblée, la procédure de notification n'a guère évolué, ce qui nous paraît plus sage. Nous considérons toutefois que l'objet du texte mériterait de bénéficier d'une navette parlementaire afin de nous permettre un temps d'analyse et de rédaction supplémentaire. C'est dans cet état d'esprit que nous attendrons le résultat des travaux de la commission mixte

eu de bonnes intuitions, entre la régulation, l'obligation de moyens et l'outil technique que vous souhaitez constituer au service de l'Arcep et du CSA pour doter notre pays d'une expertise sur ces questions.

la tentative de régulation du numérique ? Une succession de propositions de loi qui traitent de manière extrêmement ponctuelle et sectorielle des problématiques qui naissent d'un écosystème numérique

qui ne sont pas des reculs, mais qui sont vraiment minimes. Par conséquent, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous n'aurons pas fait de progrès dans la lutte contre les contenus haineux sur internet. Bien entendu, je le regrette

très particulier à toute publication ou à tout affichage ou colportage avec des infractions limitativement énumérées, un régime de prescription particulier, avec de brefs délais, ainsi qu'un régime de responsabilité en cascade. Il est évident que ce texte ne pouvait pas concerner la loi sur la liberté de la presse de 1881.